Monsieur le président, La séance est reprise. Mes chers collègues, par lettre en date de ce jour, le Gouvernement demande le retrait de l'ordre du jour du projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale et de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso, dont l'examen était prévu le mercredi 18 décembre, et l'inscription, le même jour, des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. Acte est donné de cette demande.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, après l'émouvant hommage rendu cet après-midi à nos militaires, la discussion du budget de nos armées peut paraître en décalage avec l'émotion que nous avons vécue. Ce budget traduit des moyens et sans doute une ambition, mais l'engagement de nos militaires, lui, est d'une tout autre nature et d'une tout autre essence il relève d'une certaine forme de transcendance. Je salue leur mémoire et je m'associe à la peine de leurs familles et de leurs compagnons. Madame la ministre, alors que vous avez été ces dernières heures au plus proche de ceux qui sont dans la douleur, je vous adresse toute notre sympathie. Parce que plus que jamais, notre devoir est de donner à nos troupes et au pays les moyens d'agir, abordons ce budget avec lucidité et objectivité.

La diminution des crédits du programme 212, « Soutien de la politique de défense », s'explique quant à elle par la mise en oeuvre d'une nouvelle organisation budgétaire qui se traduit par le transfert au programme 146, « Équipement des forces » des crédits de programmes majeurs d'infrastructures adossés au programme d'armement et au programme 178, « Préparation et emploi des forces » des crédits destinés aux infrastructures à caractère opérationnel. À ce stade, mes chers collègues, d'un strict point de vue budgétaire, nous ne pouvons que nous féliciter du respect de la programmation. Pour autant, ce procès ce budget traduit certaines limites et faiblesses. Celles, d'abord, de la LPM sur deux points particuliers : les autorisations d'engagement de la mission connaissent une progression très significative, de près de 20 %. Cette forte progression est une bonne nouvelle,

La mise en place d'une nouvelle politique de rémunération et d'une réforme du ministère pour en améliorer la productivité n'épuise pas l'intégralité du sujet. L'instauration de la prime de lien au service portée à hauteur de 12 millions d'euros en 2020, constitue une innovation bienvenue. Cette prime a été spécifiquement créée pour faire face à ces difficultés, même si les premiers résultats peuvent paraître contrastés. La question de la fidélisation doit inévitablement être replacée dans un contexte plus large, celui de l'amélioration générale de la condition militaire. De ce point de vue, la revalorisation indiciaire comme la réforme du système de retraite restent devant nous. deuxième point de vigilance porte sur la coopération européenne. Le système de combat aérien du futur repose sur la coopération franco-allemande. Or si la volonté politique semble au rendez-vous, le dossier est loin d'être bouclé sur le plan industriel. Le parlement allemand doit être consulté : nul doute qu'il veillera à la protection des intérêts économiques des entreprises nationales. Tout retard dans le projet aurait des conséquences graves sur la régénération de nos matériels et décalerait d'autant certains programmes comme le porte-avions qui succédera au. Par ailleurs, une approche exclusivement industrielle qui reposerait sur la seule exigence de servir les différents constructeurs conduirait à reproduire les déboires que nous avons connus avec certains hélicoptères ou l'A400M. Évoquant la coopération européenne, je ne puis passer sous silence la question plus large de nos alliances. La France est fondée à faire des propositions, et je comprends que l'on puisse s'interroger sur le positionnement de l'OTAN eu égard à une carte géopolitique en pleine mutation. Très certainement, le moment est venu pour nos partenaires européens de prendre la mesure que l'OTAN, à elle seule, n'est plus l'assurance de leur sécurité. Mais je ne suis pas certain que l'évocation de la « mort cérébrale » de l'Alliance atlantique soit le meilleur le moyen de poser le problème et de susciter leur adhésion

Je terminerai par où j'ai commencé. Parce que nous devons plus que jamais marquer notre soutien à nos armées, je vous invite, mes chers collègues, malgré les faiblesses et les réserves que j'ai pu émettre, à voter ce budget respectueux de la loi Parce que, face au drame que nos armées viennent de vivre, je ne pourrai pas comprendre que la logique budgétaire prévale sur la satisfaction des indispensables besoins de nos armées, j'en appelle à l'arbitrage du Président de la République

D'une part, 70 millions d'euros de crédits ont été annulés. D'autre part, des transferts de crédits sont une fois de plus nécessaires pour financer le surcoût des OPEX, alors que nous avions inscrit le principe du financement interministériel dans la LPM. C'est ce principe, énoncé clairement dans l'article que le Sénat a adopté en juillet 2018, qui n'a pas été respecté. Nous le regrettons. Pour ce qui concerne le programme 146, ce sont donc 167 millions d'euros qui sont consacrés au financement de ce surcoût. Ce fait nous préoccupe à l'approche de la révision de la LPM en 2021.

Nous avons suivi les discussions sur la motorisation pour laquelle il semble qu'un accord soit enfin trouvé, ce que vous pourrez peut-être nous confirmer. Une première étape est donc franchie. Cela étant, il faudra que ce partenariat, dans lequel vous vous êtes pleinement engagée, continue d'avoir le même soutien politique.

Par ailleurs, le troisième projet franco-allemand que vous aviez annoncé, le nouvel avion de patrouille maritime, semble avancer plutôt lentement. Pouvez-vous nous dire si ce dossier est sur de bons rails ? Enfin, vous le savez, nous sommes également très attachés à notre coopération avec les Britanniques dans le cadre des accords de Lancaster House, dont nous fêterons les dix ans à la fin de l'année prochaine. De quelles pistes disposez-vous, madame la ministre, pour relancer ce partenariat et envisager un Lancaster House II ?

Au-delà de ces éléments très positifs, je veux revenir sur le dossier très sensible du drone MALE- . L'idée des coopérations européennes en matière capacitaire est simple et connue en mutualisant les coûts de développement, d'une part, et en augmentant le nombre d'exemplaires produits du fait des besoins cumulés des différents pays européens participant au programme, d'autre part, on espère obtenir un matériel de meilleure qualité à un coût moindre. Évidemment, ces objectifs louables contrastent avec les difficultés inhérentes à tout partage de décision entre plusieurs pays. Les écueils sont de deux natures. « Le premier est le risque de « sur-spécification » : on finit par chercher à produire un mouton à cinq pattes. a trait à la logique industrielle, c'est-à-dire, pour parler crûment, l'absence de logique industrielle qui conduit d'abord, pour un pays, à réclamer la partie sur laquelle il est le moins compétent pour chercher à monter en gamme et acquérir une compétence. Ensuite, il y a la logique de retour géographique qui consiste

Notre inquiétude est que, à ce prix-là, les États participant au programme n'achètent pas, ou pas dans les quantités promises, sans même parler des perspectives d'exportation, qui seraient compromises si le prix se La tentation peut alors exister, même pour les pays qui ont participé à ce programme, d'acquérir un matériel non européen ou, du moins, d'acheter un vecteur sur étagère pour y greffer une charge nationale.

Il faut souhaiter que ce dossier puisse évoluer favorablement, car, rappelons-le, l'Eurodrone doit être l'une des composantes du SCAF. C'est pourquoi nous souhaitons vous faire part de notre préoccupation et recueillir votre analyse actuelle sur le sujet. » La parole

La nuance, légère, concerne les crédits pour les études amont : certes, ceux-ci progresseront de 62,5 millions d'euros pour s'établir à 821 millions d'euros, mais cette progression est légèrement inférieure à ce qui était prévu dans la loi 2018. On attendait en effet à l'époque 832 millions de crédits pour les études amont en 2020. Vous vous souvenez, madame la ministre, que nous avions justement souhaité inscrire cette

d'autre part, nous entendons dire que l'Onera, contrairement aux années précédentes, ne serait plus exempté de la mise en réserve de crédits, ce qui diminuerait encore son budget disponible de 2 millions d'euros.

Rappelons que, dans le même temps, le budget de l'équivalent allemand de l'Onera progresse régulièrement. Il est passé de 130 millions d'euros au début de la décennie à 180 millions d'euros

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le niveau des menaces n'a pas diminué, comme nous en avons fait le constat au début de la semaine dernière. Il justifie les efforts entrepris dans le domaine du renseignement.

Pour la DGSE, cette hausse concerne principalement les grands programmes interministériels et la cyberdéfense, qui font également l'objet, en cours d'exercice, de transferts de crédits complémentaires des services du Premier ministre et des armées. En effet, la France ne s'est pas dotée d'un service technique de renseignement comme la (NSA) aux États-Unis ou le (GCHQ) en Grande-Bretagne. Les grands programmes sont développés par la direction technique de la DGSE au profit de l'ensemble de la communauté du renseignement, et certaines capacités cyber sont partagées avec les armées. Il est donc logique que le financement de ces programmes soit mutualisé. Pour la DRSD, l'enjeu est de renforcer les capacités, tant pour la mise en oeuvre des missions de contre-ingérence que pour la détection et la réduction des vulnérabilités dans le secteur de la défense.

Les effectifs de la DGSE comme de la DRSD progressent conformément aux prévisions de la loi de programmation militaire. Grâce aux dispositions prises, tant pour améliorer la communication et le recrutement que pour fidéliser certains agents, y compris à travers un assouplissement des règles de rémunération, en 2020, la DRSD devrait combler l'important retard accumulé par rapport à son schéma d'emplois.

Au-delà des rémunérations, le problème a un aspect structurel dans un certain nombre de spécialités. Il me paraît nécessaire que des politiques d'orientation et d'incitation soient mises en oeuvre pour promouvoir les filières de formation scientifique et linguistique, ce qui permettrait de réduire ces tensions. Où en êtes-vous, madame la ministre, du dialogue avec les universités et les grandes écoles ?

en ce jour si particulier pour lui et sa famille : « Le programme 178 voit ses crédits de paiement augmenter de 13,8 % par rapport à 2019 pour s'établir à 10 milliards d'euros, soit 1,21 milliard d'euros supplémentaires en crédits de paiement.

La poursuite du « resoclage » budgétaire des surcoûts des OPEX devait s'accompagner d'une hausse à due proportion de l'enveloppe globale des crédits du programme. Or tel n'est pas le cas,

L'autre facteur d'explication de la hausse du budget du programme 178 est le transfert de crédits d'infrastructures depuis le programme 212, soit 879 millions d'euros. La mise à disposition de ces crédits s'inscrit dans le cadre de la réforme visant à responsabiliser les commandements, qui seront en mesure de prioriser leurs besoins. Cette réforme redonne globalement des leviers aux commandants des bases de défense et aux armées sans pour autant remettre en question les structures organisationnelles des soutiens dont la « militarité » est réaffirmée pour restaurer la cohérence organique des armées. « La contraction des crédits alloués à l'entretien programmé du matériel pour 2020 est surprenante au vu des résultats décevants en termes de disponibilité technique opérationnelle. La verticalisation et la globalisation des marchés d'entretien des équipements aéronautiques constituent un changement de pratique qui ne fonctionnera que si la performance est au rendez-vous. « Il conviendra également de veiller au maintien des compétences en régie de l'État

de la durée de mise en oeuvre des contrats opérationnels est non plus un risque, mais une réalité. L'actualisation de 2021 doit être le grand rendez-vous de la préparation opérationnelle. Des objectifs annuels d'évolution devront être fixés selon l'article 7 de la loi de programmation militaire. Nous y serons très attentifs. Enfin, la commission s'inquiète de la consolidation des services de soutien,

ans à un an de l'ancienneté requise des infirmiers menant les entretiens préparant les dons du sang et l'aménagement des conditions de dépôt d'urgence du plasma lyophilisé universel.

principalement en raison de la sous-réalisation des cibles d'effectifs liée à un nombre de départs plus important que prévu et à des difficultés de recrutement. Ces problèmes nous préoccupent, car ils compromettent l'effectivité de la remontée en puissance affichée par la loi Pour corriger cette sous-consommation, des mesures d'ordre technique et organisationnel ont été prises. Ainsi, les modèles de valorisation des crédits de titre 2 ont été actualisés, afin de tendre vers des prévisions de dépenses plus faciles Par ailleurs, le directeur des ressources humaines du ministère des armées a été désigné comme seul responsable de programme, pour permettre un meilleur pilotage de la masse salariale. Dans le même temps, l'attractivité mobilise tous les efforts de la politique des ressources humaines avec des mesures budgétaires, notamment la prime de lien au service, une attention portée au parcours professionnel et à l'intérêt du métier, la recherche d'une meilleure conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée, en particulier à travers la mise en oeuvre du plan Famille, sans oublier la politique de reconversion. Ces efforts doivent être poursuivis et amplifiés. C'est d'autant plus nécessaire que les projets de réforme de la nouvelle politique de rémunération des militaires et des retraites suscitent des inquiétudes. La seconde préoccupation sur laquelle je souhaite insister concerne l'incidence du projet du service national universel sur le programme 212. En 2019, les armées ont été sollicitées dans le cadre de l'expérimentation conduite dans treize départements au profit de 2 000 jeunes. Au titre de la phase 1, qui correspond à un séjour de cohésion de deux semaines en internat, elles ont fourni de l'appui et du conseil, aidé au recrutement des cadres, formé les directeurs de centres et les cadres de compagnie. Enfin, elles ont conçu et animé un module consacré à la défense et à la mémoire nationales. Elles ont aussi contribué à la phase 2, en proposant des missions d'intérêt général sur le modèle des préparations militaires. Au total, en 2019, trois équivalents temps plein auront été mobilisés. Pour 2020, avec l'extension de l'expérimentation à 20 000 jeunes, l'impact sur les effectifs des armées est évalué à une vingtaine d'emplois. Si cet effort peut sembler raisonnable, il faut noter qu'aucun crédit supplémentaire n'est envisagé pour le financer, en contradiction avec ce que prévoit la loi Et nous sommes inquiets pour la suite. En effet, en cas de généralisation, la demande adressée aux armées pour la formation des cadres va mécaniquement augmenter. Qu'il s'agisse de la phase 1 ou de la phase 2, on peut craindre que les armées ne soient davantage sollicitées compte tenu de l'offre structurée qu'elles sont seules à même de produire, en cas de défaillance des autres acteurs. Qu'il s'agisse du pilotage, du statut et de la qualité des cadres, de l'organisation, de la logistique et des capacités d'accueil, les échos que nous avons recueillis jusqu'à présent donnent le sentiment d'un dispositif qui avance à tâtons. Il est fragile et n'est pas taillé pour passer le cap de la généralisation. De plus, les prévisions budgétaires me paraissent sous-estimées.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je concentrerai mon propos sur la politique immobilière

la proposition des associations professionnelles de militaires qui défendent un projet pour le Val-de-Grâce, lequel mériterait d'être considéré. Cela étant, le bâtiment pourrait être

plutôt que dans nos départements respectifs. Mes

le tragique accident survenu au Mali, le 25 novembre dernier, et l'hommage national que nous avons rendu aujourd'hui à nos soldats morts pour la France nous rappellent la cruauté du monde dans lequel nous vivons et l'adversité à laquelle doivent faire face nos militaires. Mon groupe s'incline devant le courage de ces hommes et face à la douleur des familles qui ont perdu un être cher. Que ce soit dans la bande sahélo-saharienne, au Levant ou ailleurs, les crises se multiplient à l'échelle internationale, leur intensité va croissante et leur nature même évolue. Madame la ministre, les échanges que nous avons eus à l'occasion du Forum de Dakar ont tous sans exception rappelé la nécessité de notre engagement au Mali, comme, plus généralement, en Afrique de l'Ouest. En outre, sur notre territoire, la menace terroriste demeure prégnante et ne saurait souffrir le moindre relâchement. Dans ce contexte, le niveau d'engagement de nos armées est particulièrement soutenu depuis plusieurs années et ne devrait pas être amené à fléchir. Répondant à ces besoins importants et croissants, fidèle à la trajectoire budgétaire tracée par la loi de programmation militaire, le budget que nous examinons aujourd'hui est au rendez-vous des engagements qui ont été pris, et nous ne pouvons, madame la ministre, que saluer votre détermination. Ce budget prévoit, en effet, une augmentation de 1,7 milliard d'euros des moyens accordés à la défense, avec des crédits de paiement en hausse de 4,5 %, s'établissant à 37,5 milliards d'euros. C'est pour nous une grande satisfaction Nous nous félicitons que ce budget de remontée en puissance et de modernisation permette tout d'abord de continuer le renouvellement des capacités opérationnelles de nos armées. Je pense à la livraison, prévue en 2020, d'un sous-marin d'attaque de nouvelle génération, le Suffren, blindés Griffon, de 4 blindés Jaguar, ou encore d'un avion ravitailleur MRTT supplémentaire. Cette arrivée de matériels témoigne des efforts et des progrès effectués en termes d'innovation. Nous en avions besoin Cet accent mis sur l'innovation se traduit également par la prise en compte des nouveaux champs de conflictualité que sont le cyber, l'intelligence artificielle et le renseignement. L'affectation dans ces domaines de 300 postes créés cette année et les 821 millions d'euros spécifiquement dédiés aux crédits d'études amont, afin de concevoir de nouvelles technologies adaptées aux conflits futurs, en attestent. Par ailleurs, ce budget pour 2020 est tout particulièrement remarquable par son effort de sincérisation, l'inscription, au titre des crédits alloués aux missions intérieures et aux opérations extérieures, d'un montant de 1,1 milliard d'euros, contre 850 millions en 2019. Cela permettra, notamment, une amélioration dans l'exécution des crédits votés, ainsi que des débats plus apaisés, nous l'espérons, sur la fin d'exécution budgétaire. Restons néanmoins vigilants, car le coût des OPEX pour les crédits du programme 178 demeure sous-évalué à ce jour. La question de la prise en charge de l'intégralité des surcoûts risque donc encore de se poser.

Vous aurez compris, madame la ministre, la satisfaction que nous ressentons à la lecture de ce budget. Mais, vous le savez, nous sommes d'éternels insatisfaits ... J'attirerai donc votre attention sur quelques points de vigilance. Le premier point concerne le maintien en condition opérationnelle des matériels et la préparation opérationnelle. En effet, le niveau de sollicitation de certains équipements au cours de ces dernières années a été bien supérieur à ce que prévoyaient les contrats opérationnels. De plus, la technologie de nos équipements modernes nécessite une main-d'oeuvre et des infrastructures bien plus coûteuses que celles de nos équipements précédents. En conséquence, la disponibilité technique opérationnelle et, plus encore, la disponibilité technique de nos matériels ont dangereusement chuté, et ce dans les trois armées. Ce fait pose de lourds problèmes pour les entraînements ou les déploiements d'urgence, avec un risque de baisse de qualité de nos forces. Nous nous inquiétons donc de voir les crédits alloués à l'entretien programmé des matériels diminuer de 3,72 %. C'est pour le moins un mauvais signal

Ces entraînements constituent un pilier des compétences, de l'efficacité et de la sécurité des personnels. Ils restent pourtant inférieurs, de près de 10 %, aux objectifs fixés. et la préparation opérationnelle de nos forces sont trop importants pour que cette situation se pérennise. Il nous semble primordial d'accorder davantage d'attention à ces sujets, afin de préserver la capacité de nos armées à répondre aux sollicitations futures, sur des théâtres d'opérations toujours plus nombreux. Le deuxième point concerne la fidélisation de nos forces. Plusieurs chantiers déterminants restent à achever, concernant la qualité du soutien santé, la politique de rémunération, ou encore la réforme des retraites. Le plan Famille, lancé voilà deux ans, dont les crédits représentent 80 millions d'euros pour l'année à venir, est également essentiel à cette démarche de fidélisation. Si certaines de ces mesures sont perçues de façon très positive par les militaires- je pense au déploiement du wifi en garnison ou à la facilitation des démarches de déménagement des avis plus contrastés ont été exprimés sur la situation du logement et les conditions d'hébergement dans les enceintes militaires, dont l'amélioration se fait quelque peu attendre. enfin, concerne la coopération avec nos partenaires européens. Alors qu'approche le dixième anniversaire des accords de Lancaster House, le contexte encore flou du Brexit chez nos voisins britanniques rend crucial le besoin de réaffirmer et d'entretenir une coopération bilatérale solide et une capacité à travailler en interopérabilité. Le projet du SCAF conduit avec l'Allemagne connaît des avancées, mais il doit cependant toujours faire face à d'importants obstacles, notamment industriels. Des divergences essentielles existent à propos de la propriété intellectuelle, ou encore du choix des motoristes. Au vu de l'importance d'une telle entreprise, espérons que ces obstacles seront rapidement surmontés. Ces remarques se veulent constructives, madame la ministre. Elles ne sauraient remettre en cause le soutien que nous vous apportons sur ce budget pour 2020. Ainsi, en ce jour anniversaire de la bataille d'Austerlitz, le groupe Union Centriste votera unanimement les crédits de la mission « Défense ». La parole

de nos soldats viennent de payer de leur vie leur engagement au service de la France. Comme tous les Français, je m'associe à l'hommage rendu à ces hommes, dont la disparation touche la communauté nationale. Ces disparitions ont rappelé, ô combien cruellement, les dangers et les risques de l'engagement de nos forces militaires sur les théâtres extérieurs, dans une lutte de chaque instant contre le terrorisme. Comme vous, j'ai entendu les voix discordantes de bonnes âmes qui s'interrogent sur la présence de la France au Mali. J'ose le dire aujourd'hui fermement : elles ne sont pas les bienvenues La France ne se bat pas simplement pour le Mali ; elle se bat pour la sécurité d'une région entière et, au-delà, pour celle de notre pays et de l'Europe. J'entends être clair : ce serait une étrange manière de lutter contre le terrorisme de vouloir aujourd'hui se retirer de ce territoire et d'offrir ainsi une base aux terroristes ! La sécurité des Français et des Européens, ce n'est pas de la poudre de perlimpinpin ... S'il me paraît difficile de remettre en cause l'opportunité stratégique de l'opération Barkhane, pour autant,

En premier lieu, il est nécessaire d'amener enfin les pays européens à s'engager à nos côtés, pour notre sécurité commune. Nous entendons, de-ci de-là, bien des commentaires sur notre isolement au Mali. C'est, osons le dire, faire peu de cas des opérations de formation de l'armée malienne menées par l'Union européenne depuis 2013, ou encore du soutien américain en termes de renseignement grâce aux drones Reaper. Reconnaissons néanmoins que, dans les opérations de combat, la France reste, hélas, le seul pays occidental qui se retrouve véritablement sur le terrain. Aussi, madame la ministre, nous vous encourageons à accentuer vos efforts pour bâtir une coalition des forces spéciales européennes. En second lieu, pour coller à la discussion budgétaire qui nous réunit, il convient de s'interroger sur l'adaptation de notre armée sur le plan opérationnel au profil de l'ennemi qui nous préoccupe désormais, le combattant menant une guerre « asymétrique Dans ce cadre, et pour l'armée de terre, nous attendons le plan stratégique qui devrait tirer les conséquences de l'évolution de ces interventions. J'ose espérer qu'il nous sera présenté l'année prochaine, conformément au calendrier annoncé Ce qui est certain, c'est que face à des organisations armées qui s'adaptent et font preuve d'une agressivité sans cesse renouvelée il faudra sans cesse nous réinventer. L'intensité des interventions- je pense plus particulièrement aux OPEX -soulève moult questions, et je fais mienne cette formule, datant de 2017, du général François Lecointre, chef d'état-major des armées : « L'armée française avait été une armée de non-emploi pendant toute la guerre froide, elle est devenue une armée d'emploi, elle est même une armée extrêmement employée ». Trop peut-être, au regard des moyens dont elle disposait L'effort budgétaire consenti pour la défense doit être à la hauteur des enjeux stratégiques d'aujourd'hui. C'est chose faite, puisque le budget pour 2020 de la mission « Défense » s'inscrit dans la trajectoire fixée par la dernière loi de programmation militaire, avec 1,7 milliard d'euros de crédits supplémentaires par rapport à 2019. Je salue la poursuite des commandes et livraisons qui devaient garantir la modernisation de notre armée : les blindés Griffon, très attendus, ou encore le sous-marin Suffren, un exemple d'excellence technologique. Pour autant, j'ai souhaité reprendre quelques-unes des observations des rapporteurs. Il s'agit, d'abord, de la baisse de 3,72 % des crédits de paiement d'entretien

Vous rappelez régulièrement que nous sommes face à un budget à hauteur d'homme, et près de 80 millions d'euros seront affectés au plan Famille, contre 57 millions d'euros Toutefois, ces efforts sont-ils à la hauteur des sacrifices que nous demandons à ces femmes et à ces hommes qui se battent pour nos valeurs, pour la démocratie, pour la France et pour l'Europe ? Il importe, en ces temps de doute, d'incertitude et d'inquiétude, de ne pas relâcher l'effort sur la ressource humaine, qui, en l'occurrence, est le nerf de la guerre Si l'actualité démontre parfois avec gravité ce que signifie l'engagement, elle rappelle aussi, avec ces drames, le courage et le dévouement de celles et de ceux qui servent notre pays. Ces réserves exprimées, madame la ministre, mes chers collègues, et parce que la mission va dans le bon sens, celui d'un accroissement constant des moyens accordés à nos armées, le

Aujourd'hui même, la Nation tout entière a rendu hommage à ses héros. Treize soldats français morts pour la France, dans la lutte sans merci que notre patrie mène contre le terrorisme, au nom de la liberté et de la paix. familles meurtries, pour lesquelles nous ne cesserons d'avoir une pensée émue et parmi lesquelles se trouve celle de notre collègue Jean-Marie Bockel. Notre mémoire demeurera intacte. Face au sacrifice et à l'abnégation de nos soldats, face à leur immense courage, aucun mot ne saurait exprimer la profonde reconnaissance qui est la nôtre. Nous leur devons le respect. C'est au nom de ce sacrifice que nous, élus de la Nation, devons soutenir le combat qu'ils mènent sans relâche contre l'obscurantisme menaçant nos libertés et la paix. Notre devoir est de relayer le sens de la mission Barkhane, de ce combat contre le terrorisme au Sahel que nous devons poursuivre. Comme vous l'aviez affirmé, madame la ministre, ce combat « appartient au temps long Le Mali et le Sahel, en général, sont la proche frontière du sud de l'Europe. Les groupes armés terroristes qui sévissent dans la région déstabilisent les États du Sahel, affaiblissent les autorités locales, usent de la propagande pour délégitimer les opérations militaires internationales sur place, s'en prennent aux militaires déployés et intimident les populations civiles. Dans cette région grande comme l'Europe, ils créent des zones de non-droit qui menacent notre propre sécurité. Nous nous battons donc pour que le Sahel ne devienne jamais un sanctuaire terroriste à notre porte. Avec les Britanniques, les Danois, les Espagnols, les Estoniens, les Belges, et bientôt les Tchèques, nous nous battons pour garantir la sécurité du territoire européen. Comme vous, madame la ministre, nous sommes convaincus qu'un sursaut de la part de nos autres partenaires européens est nécessaire, et qu'il est de leur intérêt d'unir nos forces au Sahel. Ce sujet ne manquera pas d'être évoqué demain, à Londres, à l'occasion du sommet exceptionnel de l'OTAN. Madame la ministre, devant la Haute Assemblée, vous avez appelé les pays européens à constituer, ensemble, un pilier au sein de cette organisation. Vous avez raison Nous vivons un moment crucial. La crise profonde que traverse l'OTAN entache la force de la solidarité et de l'unité entre alliés. Elle nous oblige à réfléchir ensemble sur le sens et l'avenir de l'Alliance atlantique, sur la force stratégique de nos engagements et, plus largement, sur l'architecture sécuritaire de notre continent. Monsieur le président de la commission des affaires étrangères, vous avez eu les mots justes, vendredi dernier, lorsque vous avez présenté la photographie de l'état instable du monde d'aujourd'hui et évoqué le nécessaire « réveil stratégique de l'Europe, qui doit apprendre à se défendre seule Je reprends donc vos paroles, qui résument parfaitement les enjeux de ce sommet à Londres : « il faut utiliser le moment de crise que nous vivons pour aller vers une Europe plus forte dans une OTAN plus forte Pour cela, il est urgent de travailler à la redynamisation des fondamentaux de l'Alliance atlantique et, simultanément, à l'autonomie stratégique européenne et au développement d'une véritable culture stratégique commune, tout en consolidant l'industrie de défense européenne. Nous ne pouvons donc que soutenir l'action en ce sens du Président de la République, demain à Londres, où un autre dossier brûlant sera d'ailleurs discuté, celui de l'offensive turque dans le nord-est syrien. offensive, qui est venue saper des années d'efforts en matière de lutte contre le terrorisme, a ébranlé, encore une fois, la maison otanienne. Dans ce contexte géopolitique des plus tendus et des plus incertains, ce budget de la défense pour 2020 est, à la fois, équilibré et ambitieux. Il envoie un message de crédibilité politique à nos partenaires. Il atteint 37,5 milliards d'euros à périmètre constant, ce qui représente un effort national de défense de 1,86 % du PIB et une hausse de 4,5 % par rapport à 2019. C'est un budget des engagements tenus, puisqu'il est en tout point conforme à la trajectoire établie lors de la loi de programmation militaire pour les années 2019 à 2025. Dans cette deuxième année de mise en oeuvre de cette loi, un effort particulier est consenti en faveur d'un modèle d'armée « à hauteur d'homme Le renforcement des équipements d'accompagnement et de protection des soldats se poursuit, à travers le déploiement du programme Combattant 2020 et une hausse de 150 millions d'euros des crédits dédiés. Ainsi, en 2020, la totalité des militaires déployés en OPEX seront dotés du nouveau treillis et du gilet pare-balles nouvelle génération. Le plan Famille lancé en 2018 se poursuivra aussi, et 80 millions d'euros lui seront consacrés. Plusieurs mesures d'action sociale et de reconversion sont prévues. De plus, ce budget confirme la priorité accordée à la remise à niveau des hébergements au sein d'enceintes militaires, avec un plan Hébergement de 120 millions d'euros, ainsi que 540 millions d'euros pour la maintenance et l'entretien des infrastructures. Alors que se prépare le chantier de la nouvelle politique de rémunération des militaires, ce budget consacre 40 millions d'euros à l'amélioration de la fidélisation des personnels et de l'attractivité des carrières du ministère. On y trouve notamment la nouvelle prime de lien au service. Ensuite, avec 14,7 milliards d'euros de crédits d'engagement et 6,8 milliards d'euros de crédits de paiement, le budget en forte hausse alloué aux équipements se traduit par du matériel adapté aux besoins de nos armées et au meilleur niveau technologique, comme ce sera le cas avec la livraison du premier sous-marin nucléaire d'attaque, le Suffren, ou encore la poursuite du déploiement du programme Scorpion pour l'armée de terre. Enfin, nous nous félicitons que, pour la première fois, la dotation initiale prévue au titre des OPEX passe à 1,1 milliard d'euros, conformément à la loi de programmation militaire.

et sécurisé. Je conclurai en saluant, madame la ministre, votre engagement infaillible auprès de nos armées. Parce que ce budget est ambitieux, qu'il prépare notre défense de demain et qu'il garantit notre autonomie stratégique, le groupe La République En Marche votera avec conviction

nous pensons aussi aux 30 000 hommes et femmes qui sont déployés en opération, sur le territoire national comme à l'extérieur. J'aime cette pensée de Thucydide, rappelée par le général Lecointre : « La force de la cité ne réside ni dans ses remparts ni dans ses vaisseaux, mais dans le caractère de ses citoyens ». Nous mesurons pleinement aujourd'hui, par la dignité des familles et des frères d'armes endeuillés, la justesse d'une telle affirmation. Oui, mes chers collègues, l'excellence de nos armées provient surtout de la qualité des femmes et des hommes qui les servent : aviateurs, marins, soldats, qui ont en partage les valeurs militaires de respect, d'abnégation, de solidarité, de courage, valeurs qui irriguent et fortifient l'ensemble de la Nation. Dans un monde « ensauvagé » par des crises toujours plus nombreuses et plus violentes, pour voir clair dans le brouillard de la guerre, dans la poussière des conflits, des guérillas, face à la brutalité du terrorisme, nos forces armées sont un rempart et une boussole.

L'effort sur la condition du personnel et les infrastructures se poursuit. Les problèmes d'attractivité et de fidélisation, bien que non entièrement résolus, sont pris en compte. Tout n'est pas parfait, mais nous sommes vraiment sur une bonne trajectoire, et je veux à mon tour, madame la ministre, vous rendre hommage et saluer votre détermination sans faille et votre pugnacité pour obtenir ces résultats.

un bémol doit être apporté : 70 millions d'euros ont été annulés dans le collectif sur la mission « Défense ». En outre, pour le financement du surcoût des OPEX, le Gouvernement a pratiqué la solidarité ministérielle inversée.

dans le contrat, qu'en sera-t-il lorsque nous en serons à la seconde partie de la loi de programmation militaire, à partir de 2022, avec des marches aussi redoutables que 3 milliards d'euros d'augmentation de crédits chaque année ?

! Nous, les politiques, nous leur devons le respect de la parole donnée ! C'est une véritable question de confiance ! C'est pourquoi, encore une fois, nous souhaitons vous soutenir dans vos efforts pour maintenir le cap de ce budget,

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, tout d'abord, je souhaite à mon tour rendre hommage à tous nos soldats tombés en opération. Engagés pour notre sécurité et notre liberté, volontaires pour toutes les missions au service de la paix, ils font preuve d'un courage remarquable. Nous ne le dirons jamais assez, ils font la fierté des Français et l'honneur de la France. J'ai, en cet instant, une pensée particulière pour notre collègue et ami, ancien ministre, Jean-Marie Bockel, lui-même membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Nous lui présentons, ainsi qu'à sa femme et à ses proches, nos plus sincères condoléances. Nous pensons à son fils et aux douze camarades de celui-ci, tous disparus au Mali. Nous pensons à eux, et à tous les autres Nos soldats sont de grands professionnels, formés au plus haut niveau et parfaitement encadrés. J'ai pu le mesurer dans mes précédentes fonctions, chaque fois que j'ai eu l'honneur de leur rendre visite. J'ai pu observer le travail quotidien d'entraînement, la constance de la pédagogie, la répétition inlassable des techniques, le savoir-faire incroyable dans les déploiements opérationnels, l'évaluation permanente des risques, l'apport décisif de nos renseignements Toutes ces dispositions conduisent à des décisions d'engagement en conscience. Je peux en témoigner : tout est mis en oeuvre, afin que les femmes et les hommes composant nos armées prennent le moins de risque possible. Tout est mis en oeuvre pour qu'ils puissent réaliser leur mission au service de la patrie. Malheureusement, nous le mesurons comme eux-mêmes, toutes les missions qui leur sont confiées comportent leur part de risques. C'est en conscience que nos militaires s'engagent au péril de leur vie. est la grandeur de leur service. Personne ne peut douter de leurs principes et de leurs valeurs. Nos soldats « serv[ent], sans se servir ni s'asservir », portant le devoir avant tout.

dont le courage est quotidien et dont la force mentale est exceptionnelle, quand leurs forces physiques s'amenuisent. Ils se relèvent, appuyés par les personnels du service de santé des armées et de l'Institution nationale des Invalides. Ils se relèvent grâce à la présence, à leurs côtés, de leurs familles et de leurs camarades, qui ne laissent jamais personne derrière eux. En pensant à nos soldats, nous admirons la solidarité et les liens de fraternité qui les unissent, des liens solides et durables, exemplaires pour l'ensemble de notre société. La professionnalisation des armées a, de ce point de vue, largement renforcé cette unité en rapprochant encore plus les chefs de leurs troupes. J'ai pu m'en rendre compte à de nombreuses occasions, notamment lorsque j'ai eu à passer les fêtes de fin d'années à leurs côtés, ou au cours de mes échanges avec les différents chefs d'état-major. Madame la ministre, nous examinons aujourd'hui les crédits de la mission « Défense », dans le cadre du projet de loi de finances pour l'année 2020.

Votre collègue ministre des affaires étrangères sera heureux de l'apprendre. Nous saluons l'augmentation des crédits de 1,6 milliard d'euros, portant le budget à plus de 37 milliards d'euros pour 2020. Cette hausse place l'effort à hauteur de 1,86 % du PIB, et la trajectoire vers l'objectif de 2 % en 2025 semble respectée, telle qu'elle est précisée par la LPM. En matière de budget pour la défense, nous remarquons que le gouvernement actuel poursuit le travail engagé dès 2012, sous la présidence de François Hollande. Ce budget comporte de véritables avancées en termes d'équipements, avec les livraisons attendues de 12 000 fusils HK416F, qui complètent le remplacement des Famas, de 128 Griffon, ou encore des hélicoptères NH90, des deux A400M Atlas ou des deux premiers Mirage 2000D rénovés. Entre autres avancées, figurent aussi le plan Famille, avec 80millions d'euros, et les 120 millions d'euros affectés à l'hébergement des militaires et de leurs familles. Nous pouvons aussi saluer le recrutement de 300 ETPT dans le renseignement et la cyberdéfense. Néanmoins, si nous saluons de manière générale ce budget et si nous voterons en conséquence, nous souhaitons aussi vous faire part de nos nombreuses interrogations. le recrutement et la fidélisation des personnels, nous sommes toujours en attente de la présentation d'un véritable plan de recrutement de hauts potentiels pour nos services de renseignement et de cyberdéfense.

Les formes de l'engagement ont changé pour nos jeunes soldats. Comment prendre ce fait en compte ? Quelles sont les perspectives au-delà de l'actuel plan Famille, qui, à bien des égards, est un plan de rattrapage, dans la continuité des rattrapages déjà effectués lors du précédent quinquennat ?

À l'heure où nous parlons, plus de 30 000 militaires sont engagés pour la défense de la France : parmi eux, 8 000 sont en OPEX, pour l'essentiel dans la bande sahélo-saharienne et au Levant 20 000 sont engagés sur le territoire national, dans le cadre des postures permanentes de sauvegarde maritime ou de sûreté aérienne, dans l'opération Sentinelle, au sein de nos forces de souveraineté dans nos collectivités d'outre-mer 3 700 sont prépositionnés comme forces de présence à l'étranger. Comme le dit le général Lecointre : « rapporté à nos effectifs aujourd'hui, ce niveau d'engagement soutenu depuis de nombreuses années est inédit et il ne devrait pas fléchir dans les années à venir ». Nous ne pouvons que partager le constat et les observations du chef d'état-major des armées. Malheureusement, si ce budget est en augmentation et apparaît comme une réponse à court et peut-être moyen termes, il ne semble pas, ou pas encore, répondre aux enjeux à long terme. Vous paraissez en avoir conscience, madame la ministre, puisque vous avez posé peu ou prou le même constat, lors d'une conférence que vous avez donnée en septembre dernier. Les guerres de demain appellent des décisions aujourd'hui.

La compétition est déjà lancée. La France n'est pas complètement sortie du jeu, mais elle connaît des retards significatifs, dans un environnement sécuritaire où ses forces sont fortement mobilisées. L'équation est certes complexe, mais, nous le savons, ce ne sont pas les effets d'annonce et de communication qui feront que notre pays pourra se défendre face à des attaques hybrides, multiples et parfois insaisissables. Dans le domaine de la défense spatiale, une réorganisation a été annoncée et fortement commentée. Elle est en cours, mais des investissements réels et pérennes dans ce secteur encore largement inexploré ? Voilà un défi redoutable gérer le quotidien de nos armées tout en les projetant vers l'avenir. L'Europe de la défense semble la seule hypothèse solide et durable, mais, là encore, nous notons des annonces régulières et largement partagées, mais peu d'avancées concrètes. Nous avons conscience des difficultés de cette équation à plusieurs inconnues, dans un environnement mondial en permanente mutation. Nos concitoyens, et parmi eux nos soldats, attendent aussi des réponses concrètes sur le long terme.

Pour autant, cela ne nous empêche pas de constater et de relever tous les effets négatifs d'un mauvais projet de loi de finances pour l'année 2020, qui enrichira encore plus les très riches sans redistribuer réellement à celles et ceux de nos compatriotes qui en ont le plus besoin, plus besoin, dans un climat social terriblement effrayant pour la plupart des Français, qui s'inquiètent, quel que soit leur niveau au sein de notre société, des étudiants aux familles, des salariés aux entrepreneurs, de nos jeunes à nos anciens. Le groupe socialiste continuera à dire son opposition entière à la politique économique et sociale du gouvernement actuel ; cependant, il votera les crédits de la mission « Défense ». Nous le devons à nos militaires, à leurs familles et à nos concitoyens

L'hommage national rendu aujourd'hui a honoré leur mémoire, et nous renouvelons notre soutien aux familles durement éprouvées, à notre collègue Jean-Marie Bockel, et à tous les compagnons d'armes de ces défunts soldats qui accomplissent leur mission dans des conditions chaque jour plus périlleuses. Oui, chaque jour plus périlleuses, car plus de 40 militaires français ont trouvé la mort dans la région. Nous y déployons 4 500 militaires. Outre nos forces, des soldats maliens, burkinabés, nigérians subissent des pertes plus nombreuses encore.

». Le bilan humain de cette guerre, que les populations de la région considèrent de moins en moins comme la leur, s'alourdit dramatiquement, sans que l'on voie poindre d'issue positive. Le risque d'enlisement et d'un rejet croissant des troupes françaises est maintenant manifeste. Voilà qui conduit à s'interroger sur le budget que nous examinons. Le coût des OPEX augmente fortement. Au-delà des seules lignes budgétaires directement imputées à ces opérations, une part de plus en plus importante de nos crédits d'équipement, eux aussi en forte hausse, vise en fait à accroître notre capacité de projection extérieure. N'est-il pas temps de réévaluer le bilan de cette politique, aujourd'hui au Sahel, hier en Libye, ou ailleurs encore en Afrique ou au Moyen-Orient ? Au Sahel, notre engagement est maximal ; la situation sociale, humanitaire et sanitaire se dégrade au rythme du délitement des États et de leurs politiques publiques, dû à des années d'ajustement structurel, de pillage économique, de corruption d'interventionnisme militaire et politique. Les conflits internes, la violence, les trafics et le banditisme se répandent au fur et à mesure que grandissent la pauvreté et l'absence totale de

La primauté donnée à l'action militaire s'avère désormais dangereuse pour l'Afrique, pour la France et pour nos militaires. Les équilibres de notre politique extérieure en matière de développement, de diplomatie et d'action militaire doivent être revus. Quels sont-ils aujourd'hui ? Un budget militaire en hausse tourné vers l'opérabilité extérieure, une diplomatie aux moyens sans cesse rognés, et une aide au développement qui ne décolle pas malgré les promesses ... Nous marchons sur la tête Remettre notre politique à l'endroit doit nous permettre de changer nos rapports politiques et de développement avec les États et les forces vives en Afrique. C'est le seul moyen d'éviter l'enlisement, dans une guerre qui devient chaque jour plus meurtrière. plus meurtrière. Le premier de nos désaccords porte donc sur les opérations extérieures. Plus globalement, nous souhaiterions que l'augmentation des budgets consacrés à la modernisation de nos équipements soit revue à l'aune d'une révision stratégique d'ensemble. Nous ne visons pas là les conditions matérielles de nos soldats, marins et aviateurs, qui, eux aussi, ont subi de dures années d'austérité et méritent cette remise à niveau. Nous visons, par exemple, l'intégration croissante dans les stratégies de l'OTAN de nos objectifs en matière de dépenses militaires et de nos concepts d'emploi des forces, d'emploi des forces, alors même que l'Organisation est fortement remise en question. Quelles conclusions tirons-nous de ce qui vient de se passer en Syrie, avec le retournement de nos alliés ? Quel est le coût budgétaire de notre engagement dans le commandement intégré ? Depuis les propos du président Macron sur la « mort cérébrale » de l'Organisation, les déclarations gouvernementales censées les expliquer ne nous éclairent pas beaucoup sur notre vision d'avenir.

allons voter ce budget sans disposer de réponses claires à cette question pourtant essentielle. Nous visons aussi les stratégies de nos industries de défense, qui s'imbriquent progressivement en Europe, sans que des doctrines d'emploi communes, à l'exception de celles de l'OTAN, ne soient mises au clair. L'Europe de la défense ne serait-elle pas, pour le moment, qu'une Europe des industriels de la défense, dictant les programmes à financer, plutôt qu'un projet politique commun à débattre et à arbitrer avec les parlements et les citoyens ? Ces industries de défense se tournent également toujours plus vers des stratégies agressives à l'export, nourrissant un commerce des armes florissant, devenu dans ce contexte géopolitique instable l'un des principaux facteurs de dangers, de conflits et de violences.

pour défendre notre souveraineté, pour défendre notre liberté et pour défendre nos valeurs.

indispensable et nécessaire. Cela faisait trop longtemps, madame la ministre, que nous n'accordions pas les moyens nécessaires à notre défense.

chose, le départ de Donald Trump pour mettre sous le tapis cette Europe de la défense que nous avons peut-être, dans les mois à venir, la possibilité de construire. Des mutualisations existent déjà, je m'en félicite.

La mutualisation de la production a de nombreux avantages et renforce notre interdépendance. Mais elle présente l'inconvénient politique de devoir s'appuyer sur une Europe puissante, intégrée et politiquement forte.

aux proches et aux frères d'armes des treize soldats tombés au combat, au Mali, lundi dernier. Au nom du groupe Les Républicains du Sénat, je veux redire à quel point nous saluons leur courage de chaque instant et leur professionnalisme. Aujourd'hui, mais pas seulement, nos pensées les accompagnent. Face à leur engagement jusqu'au sacrifice ultime, nous devons les assurer de notre soutien indéfectible et de notre profonde compassion. La Nation doit être au rendez-vous et soudée derrière ses soldats et héros de la lutte mondiale contre le terrorisme, tant à l'étranger que sur le territoire national. Oui, la paix, ici et en Europe, se joue là-bas. Madame la ministre, le budget que vous nous soumettez respecte la trajectoire tracée par la LPM, pour laquelle nous nous sommes tous beaucoup investis. C'est donc avec satisfaction que nous constatons que, en 2020, le budget de la défense atteindra 37,6 milliards d'euros, ce qui représente une hausse de 1,7 milliard d'euros. Ce budget comporte des avancées qu'il convient de souligner. Concernant les équipements, les efforts en termes de matériel étaient très attendus. Il y va de la sécurité de nos soldats. Cette année est marquée par la poursuite de la modernisation des équipements conventionnels, avec une hausse de 1,3 milliard d'euros, qui se traduit notamment par la livraison du premier sous-marin nucléaire d'attaque de nouvelle génération, le Suffren. L'année 2020 verra également le déploiement du programme Scorpion, avec la livraison de blindés multi-rôles, tels que les Griffon. À cela s'ajoute la livraison d'un avion ravitailleur MRTT supplémentaire, permettant de renforcer nos capacités, jusque-là critiques, de ravitaillement en vol. Cette modernisation se caractérise aussi par le lancement d'études sur le sous-marin nucléaire lanceur d'engins de troisième génération, et réaffirme la crédibilité de la dissuasion nucléaire française dans ses deux composantes. Ces efforts sont indispensables pour la France, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et membre de l'OTAN. Si la livraison de nouveaux matériels est importante, l'autre chantier relatif aux équipements est celui de la mise en place d'une politique de maintien en condition opérationnelle (MCO) rénovée, intégrant les spécificités de nos opérations extérieures. Le groupe Les Républicains est très attentif à la gestion du surcoût des OPEX, qui atteint 1,1 milliard d'euros, en particulier du fait de la fin du financement interministériel. La prise en charge par la solidarité nationale a un sens ; c'est

Si nous ne voulons pas nous retrouver dans la situation des Britanniques après leurs interventions simultanées et prolongées en Afghanistan et en Irak, l'amélioration de l'efficacité du maintien en condition opérationnelle n'est pas négociable. Le rapport de Dominique de Legge relatif à la disponibilité des hélicoptères constituait un excellent exemple. La réforme engagée est un signe positif, mais la baisse de 3,72 % des crédits dédiés à l'entretien programmé du matériel ne laisse plus aucune marge de manoeuvre. Il faut donc rester extrêmement vigilant, car les conséquences sur l'activité et l'entraînement des forces sont immédiates. Le nombre d'heures d'entraînement pour les personnels est un gage autant de professionnalisme que de sécurité. Cependant, préserver nos capacités matérielles exige une politique soutenue en matière d'innovation. Les investissements en termes de recherche et développement sont le préalable indispensable à une base industrielle et technologique de défense solide et pérenne. Il importe de nous prémunir contre tout décrochage technologique, qui anéantirait les efforts consentis jusqu'à présent. À ce titre, la part relative aux études amont, le programme 144, représente un défi. Cela doit amorcer la montée en puissance de l'Agence de l'innovation de défense. Intelligence artificielle, informatique quantique, hypervélocité, cybersécurité, spatial et neurosciences sont des domaines totalement intégrés à toute politique de défense. Néanmoins, chacun est conscient qu'il ne peut y avoir de défense sans les hommes et les femmes, des soldats qui ont des familles, dont nous devons aussi nous préoccuper. Dans ce cadre, le plan Famille est un élément essentiel.

La fidélisation est un défi qu'il faudra relever. Cela ne peut s'envisager sans une amélioration de la gestion des carrières, avec une vision à long terme. Cette tâche immense exige un alignement sur les rémunérations du domaine civil. L'armée doit séduire et recruter auprès des jeunes, qui suivent un enseignement et des formations de qualité au sein de la défense. Il importe que la défense puisse avoir un retour sur cet investissement. J'en viens au service national universel (SNU), qui peut potentiellement avoir un effet sur les recrutements. Les membres de la commission des affaires étrangères seront intraitables sur le financement, qui doit faire l'objet de ressources. Il y va du respect de la loi de programmation militaire. Que l'armée prenne sa part, et seulement sa part.

Madame la ministre, le groupe Les Républicains votera les crédits de la mission « Défense ». Toutefois, ce vote favorable s'accompagne d'une extrême vigilance quant au strict respect de la loi de programmation militaire, gage du respect que nous devons à toutes les femmes et à tous les hommes engagés au service de la défense. Nous leur sommes quotidiennement reconnaissants.

pour rendre hommage à nos treize militaires morts pour la France au Mali et témoigner à leurs familles et leurs proches le soutien et la reconnaissance de la Nation tout entière. cercueils drapés de bleu, blanc, rouge, ces treize vies consacrées à notre pays et à notre protection nous rappellent que celles et ceux qui choisissent de s'engager le font corps et âme, sans retenue ; ne l'oublions jamais. je tiens à vous remercier, mesdames, messieurs les sénateurs, de votre soutien indéfectible dans cette terrible épreuve. En cette journée de deuil et d'hommage, la présente séance publique revêt une dimension particulière, parce que nous sommes au Sénat, parce que nous examinons les moyens alloués à nos armées, et parce que votre collègue et notre ami Jean-Marie Bockel aurait dû prendre la parole en tant que rapporteur pour avis Permettez-moi de lui adresser une pensée affectueuse et de lui exprimer tout notre soutien. Nous sommes réunis ce soir pour examiner le deuxième projet de loi de finances de mise en oeuvre de la loi de programmation militaire. Nous avons pris des engagements forts dans cette loi de programmation voulue par le Président de la République pour la remontée en puissance de nos armées, afin que, dans un environnement stratégique qui se dégrade chaque jour, jamais les armées ne faillissent à leur mission première : protéger les Français. Les armées ont déjà connu par le passé des LPM devenues obsolètes à peine promulguées. Cette loi de programmation militaire voulue par le Président de la République n'est pas une promesse ; c'est un cap que nous avons fixé et que nous comptons bien tenir. Pour la troisième année consécutive, le budget de la mission « Défense » est en hausse. Comme le prévoyait la loi précitée, en 2020, nous bénéficierons de 1,7 milliard d'euros de crédits supplémentaires à périmètre constant, ce qui porte notre budget à 37,5 milliards d'euros. C'est une hausse de 4,5 % par rapport à 2019, dans un contexte budgétaire contraint pour l'État. Elle marque la priorité donnée par le Gouvernement à la poursuite du renforcement des fonctions régaliennes, les armées au premier rang. C'est aussi la marque du respect de l'engagement fort du Président de la République de porter l'effort national de défense à 2 % de la richesse nationale d'ici à 2025. Cet objectif n'est pas seulement symbolique. Il est indispensable pour réparer et préparer nos armées. En outre, et c'est une chose à laquelle je tiens- je sais que vous aussi c'est un budget sincère. Il est constitué exclusivement de crédits budgétaires. La provision destinée à couvrir le surcoût des OPEX et des missions intérieures atteint désormais un niveau bien plus réaliste et sécurisé, avec 1,1 milliard d'euros cette année, auxquels s'ajoutent 100 millions d'euros pour les opérations intérieures, soit 1,2 milliard d'euros au total. d'euros -est à comparer avec la prévision de surcoûts pour 2019, soit 1,4 milliard Cela réduira encore la traditionnelle tension de la fin de gestion, que l'on a constatée par le passé, comme en 2016 ou 2017, quand la provision s'élevait à 450 millions d'euros, laissant ainsi 1 milliard d'euros à trouver sur le budget de l'État. J'en profite pour faire une incise sur les conditions de fin de gestion 2019 pour le ministère des armées,

Pour mémoire, le projet de loi de finances rectificative qui a été présenté voilà quelques semaines a prévu l'ouverture de 214 millions d'euros pour le financement des surcoûts liés aux opérations extérieures et aux missions intérieures, ainsi que des annulations à hauteur de 284 millions d'euros. Ce schéma de fin de gestion de la mission « Défense s'inscrit- cela a été rappelé -dans le contexte du financement des mesures en faveur du pouvoir d'achat décidées à la fin de l'année 2018, pour lequel le Premier ministre a demandé une réduction des dépenses de l'État de 1 milliard d'euros par rapport à la loi de finances initiale. Dans ce contexte, le ministère des armées compense en annulations en 2019 les ouvertures permettant de couvrir les surcoûts liés aux opérations extérieures et aux missions intérieures. Par ailleurs, pour contribuer à l'effort collectif, j'ai décidé la restitution au budget général d'un montant de 70 millions d'euros résultant des gains sur les négociations des contrats d'armement et du paiement de pénalités de retard par les industriels, ce qui est donc sans conséquence sur l'exécution de la LPM. Au total, les surcoûts liés aux opérations extérieures et aux missions intérieures d'un montant de 1,4 milliard d'euros sont intégralement couverts, avec des conséquences que je qualifierais d'absorbables par le ministère. On peut se désespérer de tout, mais rappelons quand même que le montant des annulations s'élève à 284 millions d'euros, c'est-à-dire 0,8 % du budget des armées,

C'est aussi l'illustration de l'effort de « sincérisation » qu'a permis la hausse des provisions de 450 millions d'euros dans la précédente LPM à 1,1 milliard d'euros en 2020. La gestion 2019 n'est pas finie, notamment concernant la réserve de précaution, c'est-à-dire les crédits qui restent gelés. Cette réserve, après les annulations du collectif, était de 420 millions d'euros. J'ai d'ores et déjà obtenu 80 millions d'euros de dégel à la fin du mois de novembre.

dont je demanderai le dégel intégral dès que les conditions d'atterrissage de la gestion de l'État seront confirmées, c'est-à-dire à la mi-décembre.

2020, selon les quatre axes de la loi de programmation militaire. Vous le savez, j'ai souhaité mettre l'humain, les civils, les militaires et leurs familles au coeur du ministère, au coeur de nos armées, au coeur de notre action.

Il disposera d'un budget d'environ 80 millions d'euros en 2020, contre 57 millions d'euros en 2019. Ce sont par exemple de nouvelles places en crèches qui seront ouvertes à Mérignac ou à Calvi. C'est encore l'extension du déploiement du wifi en garnison et l'ouverture d'espaces Atlas pour simplifier la vie quotidienne de nos militaires. Nous consacrons également 120 millions d'euros pour améliorer les conditions d'hébergement des militaires, notamment des militaires du rang de l'armée de terre, qui en ont parfois bien besoin. C'est pourquoi 540 millions d'euros iront à la maintenance et à l'entretien des bâtiments et des infrastructures. Je sais que vous êtes particulièrement vigilants Ce projet de loi de finances n'oublie personne. Nous veillons également à améliorer les conditions de travail et de vie des agents civils du ministère des armées. Au total, 300 emplois seront créés en net en 2020 pour renforcer les domaines prioritaires du ministère, à savoir le renseignement, la cyberdéfense et le numérique. n'oublie pas non plus les équipements du quotidien indispensables à nos forces. Par exemple, conformément à nos engagements, 100 % des militaires déployés en OPEX seront dotés en 2020 du nouveau treillis ignifugé, qui les protège mieux, et 12 000 nouveaux fusils HK416F seront distribués. Les petits équipements du quotidien faisaient partie des promesses de la LPM ; nous tenons Ce ne sont pas les seuls matériels vieillissants. Nous poursuivons cette année le renouvellement des capacités opérationnelles de nos armées. Ce projet de loi de finances accélère la modernisation et le renouvellement de nos équipements. Je vous en 2020, le montant des autorisations d'engagement inscrit dans le budget sera de 14,6 milliards d'euros pour les programmes à effet majeur, soit une progression de près de 85 % en un an.

l'arrivée des Griffon, 128 pour être exacte, la livraison des quatre premiers blindés Jaguar, du sous-marin Suffren, ou encore du troisième avion ravitailleur MRTT Phénix. J'ajouterai un autre chiffre parlant sur la hausse de 1,7 milliard d'euros, deux tiers seront consacrés aux programmes d'armement majeurs pour nos armées. Comme vous pouvez le constater, chacune des armées pourra ressentir les effets de la remontée en puissance portée par cette LPM. Ce budget pour la défense, c'est aussi la consolidation de notre autonomie stratégique et une contribution supplémentaire à celle de l'Europe. Nous ne perdons pas de vue la préparation aux conflits du futur et l'innovation pour que nos forces aient toujours l'avantage sur le terrain, avec 821 millions d'euros spécifiquement consacrés à l'innovation à travers les contrats et études amont pour concevoir les technologies de demain. Il s'agit d'une hausse de 8 % par rapport à 2019. 448 millions d'euros seront consacrés à développer nos capacités spatiales et renouveler nos satellites. L'effort en matière de dissuasion se poursuivra, avec 185 millions d'euros de crédits d'études amont. Et de nouveaux cybercombattants vont rejoindre les rangs ; l'objectif est d'en recruter 1 000 d'ici à 2025.

ministère est de poursuivre sa transformation, de simplifier et d'améliorer la performance de ses processus. Vous le savez, c'est un sujet qui me tient particulièrement à coeur. Je m'assure continuellement que les chantiers de transformation et de modernisation du ministère avancent dans la bonne direction. J'ai souhaité commencer par moderniser le ministère au plus près du terrain ; je vous remercie de l'avoir noté. Ainsi, les commandants de base de défense disposent aujourd'hui de plus de latitude et de moyens pour agir. Mais il fallait aussi revoir l'organisation des états-majors, des directions et des services, pour les recentrer sur leurs missions stratégiques, les faire mieux travailler ensemble, les rendre plus efficaces, et dégager des effectifs pour les redéployer sur les fonctions prioritaires. C'est en ayant cela à l'esprit que nous réduisons le nombre de strates hiérarchiques, que nous faisons en sorte de briser les silos et que nous délocalisons certains de nos services sur les territoires hors d'Île-de-France. Je suis particulièrement attachée à la qualité d'exécution des décisions que nous prenons. C'est bien sur le terrain que nos réformes prennent corps et que la loi de programmation militaire doit être mise en oeuvre.

c'est un budget au rendez-vous des engagements de la LPM 2019-2025, un budget qui accélère les investissements en matière d'équipements, qui appuie notre volonté de concevoir et déployer des mesures à hauteur d'homme et qui confirme nos ambitions. Nous allons

peuvent être fragilisées par un manque de moyens budgétaires et un sous-effectif moyen, qui se situe aux alentours de 9 %.

de 31 % par rapport à 2019 en crédits de paiement et de 43 % en autorisations d'engagement pour 2020,

telle rationalisation des implantations franciliennes de l'Onera est l'un des objectifs majeurs de l'Office dans la période à venir. Elle a été intégrée dans les objectifs du contrat d'objectifs et de performance, qui prévoit, durant sa période d'exécution, les travaux pour rassembler les équipes et les installations de Meudon et Châtillon, avec une possibilité d'implantations supplémentaires à proximité directe d'un nouveau bâtiment de l'École polytechnique et de l'École D'un montant global évalué à 160 millions d'euros pour une durée d'environ cinq ans, le projet a été autorisé en conseil d'administration extraordinaire à la Sa couverture financière est en effet assurée en grande partie par des produits de cessions immobilières sur les sites de Meudon et de Châtillon. D'ores et déjà, les communes ont fait part de leur intention de préempter les terrains, ce qui devrait faciliter et accélérer la procédure de cession. Les ventes des emprises ne pouvant être réalisées qu'en fin d'opération, le besoin en trésorerie est important. Le financement sera assuré par une avance du compte d'affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l'État » dans l'attente de la récupération des produits de cession.

Madame la ministre, je ne suis pas certain que vous ayez totalement répondu aux interrogations de M. Marseille, mais je ne suis pas le mieux placé pour le savoir. Simplement, l'année dernière, vous aviez évoqué une échéance en 2022 ; j'ai le compte rendu de nos

en construction budgétaire en cas d'incertitudes et de risques internationaux pouvant affecter le prix du pétrole. Ce mécanisme permet une sécurisation de ces crédits et leur réajustement annuel en loi de finances. Nous souhaitons revenir sur ce sujet pour deux raisons liées à l'actualité. Premièrement, la situation politique actuelle dans le golfe Persique, particulièrement instable, nécessite une attention toute particulière, en raison du fort risque de volatilité des cours. vous êtes attentive à ce sujet, madame la ministre, et que le service des essences des armées veille tout particulièrement à ce que les contrats d'approvisionnement passés permettent d'atténuer les variations de cours et de couvrir les volumes nécessaires à la préparation et à l'activité opérationnelle des forces. Nous pensons qu'il est nécessaire d'assurer une meilleure anticipation des coûts pour les armées alors que l'actualisation de l'enveloppe financière dédiée aux carburants opérationnels n'est prévue qu'en 2021, comme vous l'avez vous-même indiqué, en prenant en compte les évolutions constatées au cours des gestions 2019 et 2020. Vous avez également indiqué qu'une extension du dispositif de couverture des risques était nécessaire au regard de la volatilité des cours. Peut-être pourrez-vous nous éclairer sur ce point. Deuxièmement, début

L'amiral Prazuck a ainsi souligné que la marine nationale, tout comme ses homologues, allait se trouver en compétition avec la marine marchande sur le marché du raffinage. Selon lui, « alors lui, « alors qu'auparavant, seules les marines de l'OTAN utilisaient exclusivement du diesel léger peu soufré, produit par des usines quasiment dédiées à notre seul usage, il va désormais nous falloir partager cette capacité de production avec la marine de commerce, qui utilise du diesel marine dont le taux de soufre, jusqu'ici toléré jusqu'à 1,5 %, va devoir descendre à 0,5 %, en application d'une norme internationale, ce qui entraînera une augmentation du coût du carburant

Quel est l'avis du Gouvernement ? Les crédits de carburant opérationnels sont évidemment essentiels pour l'activité des armées et ils font l'objet d'un pilotage spécifique par l'état-major des armées.

le cours du Brent était exactement de 60 dollars aujourd'hui même. Par ailleurs, les contrats d'approvisionnement et les mécanismes de couverture qui sont mis en oeuvre par le service des essences des armées permettent de lisser le prix d'acquisition sur une longue période et d'atténuer les variations du prix des carburants facturé aux armées. Enfin, vous l'avez rappelé, l'article 5 de la LPM prévoit une clause de sauvegarde qui permet de garantir l'adéquation de l'adaptation des dépenses de carburant des forces armées. Dès lors, et à ce stade, il ne me paraît pas nécessaire d'augmenter la ligne de crédits destinée à ces carburants. Mais nous aurons nécessairement l'occasion de reparler

Cette mesure vise à renforcer le contrôle de l'action du Gouvernement, en soumettant la LPM à un avis non contraignant d'un organe indépendant. Nous espérons

pas en cause la souplesse et l'adaptation de la LPM, qui est soumise à des aléas géopolitiques parfois imprévisibles. Il s'agit d'anticiper le plus en amont possible ces aléas, tout en assurant une exécution comptable fiable de la LPM.

Au même moment, Thierry Breton, le commissaire européen français chargé de la mise en place de ce fonds, martelait pour sa part l'importance du développement d'une industrie européenne capable de disposer de technologies souveraines en matière de défense. Dès lors, qui croire ? de la défense, dont la création a été approuvée à une large majorité en avril dernier, est destiné à développer l'autonomie stratégique européenne que la France appelle de ses voeux, en finançant l'innovation stratégique dans le domaine militaire à laquelle les industriels français peuvent prétendre. C'est la première fois que l'Europe investit en faveur de sa défense au-delà de la dimension capacitaire.